L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions

l'organisation d'un marché libéralisé de l'énergie. Si nous pouvons souscrire à l'objectif affiché de renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz et le bon fonctionnement du système gazier, les mesures préconisées ne nous semblent pas aller dans le bon sens. Nous contestons ainsi que l'on puisse envisager de recourir aux enchères pour satisfaire aux obligations de stockage. Nous relevons également qu'un arrêté du 31 juillet dernier réduit à 50 % la disponibilité des stockages de sécurité situés sur le territoire national. Une telle décision engendre précisément des risques en termes de sécurité d'approvisionnement. Par ailleurs, nous regrettons que cet article tende à autoriser le financement de l'écart éventuel entre le revenu autorisé par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, et le produit des enchères par un terme tarifaire spécifique de transport mis à la charge des consommateurs. Nous craignons, avec ce mécanisme, des hausses de tarifs pour les consommateurs. cet article des éléments de libéralisation accrue qui sont des facteurs d'insécurité pour le bon fonctionnement du système gazier. Nous revendiquons au contraire la mise en place d'une maîtrise publique, seule à même de garantir sécurité d'approvisionnement et continuité du service public, l'intervention d'un opérateur national plus soucieux de la satisfaction des besoins que de l'obtention d'un retour sur investissement. Nous appelons de nos voeux la constitution d'un pôle public de l'énergie. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de cet article. l'avis de la commission que le dispositif proposé « représente une libéralisation accrue du secteur ». Or c'est véritablement tout le contraire qu'il s'agit de mettre en oeuvre ! Jusqu'à présent, le stockage du gaz était une activité non régulée, les stockeurs pratiquaient des prix libres, sans contrôle de leurs marges, malgré une situation duopolistique, le niveau des capacités de stockage souscrites s'établissait par le seul jeu de l'offre et de la demande. Ce système a montré ses limites, car il est apparu que le marché n'était pas en mesure de révéler la véritable valeur du stockage pour la collectivité. Il est donc apparu nécessaire, pour garantir notre sécurité d'approvisionnement, de basculer vers un régime prévoyant, en particulier, un revenu autorisé des stockeurs établi par la CRE, la constitution de stocks complémentaires lorsque le marché seul ne permet pas d'atteindre le volume minimal requis pour assurer la sécurité d'approvisionnement, ou encore la socialisation d'une partie des coûts du système leur couverture par les tarifs d'utilisation des réseaux acquittés par tous les consommateurs. Le tout doit conduire, par la régulation des prix, à des économies, pour l'ensemble de la collectivité, collectivité, qui pourraient atteindre jusqu'à 100 millions d'euros, selon l'estimation des trois corps d'inspection ayant remis un rapport sur le sujet. Revenu fixé par le régulateur, imposition d'obligations nouvelles, socialisation partielle des coûts : nous sommes donc très loin d'une libéralisation accrue du secteur ! L'avis de la

ont, eux, l'obligation de souscrire des capacités de stockage à ces tarifs. La régulation des opérateurs de stockage prévue dans le cadre de la réforme doit permettre un bien meilleur contrôle du coût de stockage, au bénéfice du consommateur final. Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

pour présenter l'amendement n° 2 rectifié. Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier sont fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. Le présent amendement vise à compléter la disposition votée par l'Assemblée nationale et reprise en commission par le Sénat au 5° de l'article 4. Ce paragraphe tend à insérer un article L. 421-3-1 dans le code de l'énergie, prévoyant le principe d'un délai technique de préavis de sortie du périmètre régulé régulé pour les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel n'étant plus considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz du pays par la PPE. Les impacts sociaux et industriels d'un éventuel ajustement du périmètre régulé seraient majeurs, entraînant irrémédiablement des fermetures de sites, des suppressions d'emplois locaux et de recettes fiscales, des transferts de personnel, De plus, compte tenu de la nature de ces actifs, toute fermeture de site de stockage serait irréversible, alors même que le gaz, de plus en plus produit à partir de sources renouvelables,

Dans leurs trajectoires prévisionnelles vers un décarboné, la plupart des prospectifs à long terme incluent en effet le recours au stockage gazeux souterrain -hydrogène en mélange ou pur, méthane de synthèse considérant qu'il s'agit du moyen le plus économique pour stocker et déstocker l'électricité intermittente convertie en gaz. Dans ce contexte, alors qu'une révision de la PPE est prévue à la fin de l'année 2018, soit quelques mois à peine après

Cette visibilité sur cinq ans permettra d'avoir un retour suffisant sur le succès du dispositif de régulation pour garantir la sécurité d'approvisionnement du pays, et de ne pas préempter, par des décisions irréversibles à court terme sur des actifs, son avenir énergétique. La

régulés au-delà même de cette sortie. La transition ne sera donc pas brutale : elle donnera le temps suffisant aux opérateurs pour s'adapter. Il ne semble pas opportun d'aller au-delà, sauf à limiter la capacité de pilotage de l'État, ce qui n'est pas souhaitable.

aux nécessités de la sécurité d'approvisionnement. La programmation pluriannuelle de l'énergie est un outil parfaitement adapté pour ce faire et il n'y a pas, de notre point de vue, de justification à figer dans le temps une telle liste. Toutefois, le Gouvernement est pleinement conscient qu'un délai peut être nécessaire afin qu'un opérateur de stockage puisse préparer la sortie éventuelle d'un de ses sites de stockage du périmètre de la régulation. La réforme prévoit ainsi un délai de préavis, dont il conviendra de définir la durée adéquate dans le cadre d'une concertation avec les acteurs gaziers. Un dispositif est donc déjà prévu pour offrir de la visibilité aux opérateurs de stockage. Par ailleurs, la programmation pluriannuelle de l'énergie pourra fixer, si nécessaire, des dispositions transitoires. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques. Madame Chain-Larché, l'amendement n° 2

Cet amendement vise à permettre à des fournisseurs désignés dans le cadre d'accords bilatéraux conclus par la France avec un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, de souscrire en priorité, en amont de leur mise aux enchères, des capacités de stockage. Je précise qu'un tel accord existe déjà entre la France et la Suisse.

Cette nouvelle disposition est effectivement nécessaire pour la bonne mise en application du décret n° 2009-1078 du 26 août 2009, qui porte publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et la Confédération helvétique relatif à la sécurité mutuelle d'approvisionnement en gaz naturel. Cet accord prévoit un accès pour les consommateurs suisses

Cet amendement a un double objet. La concertation sur la responsabilité du « filet de sécurité » n'étant pas achevée, il importe de ne pas préjuger de la solution qui sera retenue. C'était du reste l'intention de notre commission, mais la nouvelle rédaction proposée pour le 9°de l'article 4 lève toute ambiguïté qui pourrait subsister sur le fait que trois options sont envisageables : la constitution des stocks manquants par les opérateurs de stockage ; leur constitution par les fournisseurs de gaz naturel ; la mise en place d'un système hybride, faisant appel aux uns et aux autres. En outre, dès lors que la nouvelle obligation pourrait être imposée aux fournisseurs, acteurs qui ne sont pas régulés, il y a lieu de prévoir des modalités de sanction. Tel est l'objet du II du présent amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Cet amendement vise à permettre la création et la réglementation de stocks stratégiques gaziers sur une partie des stockages existants, afin de couvrir des situations de crise géopolitique ou de risque climatique exceptionnel, risque qui s'est déjà réalisé. En s'assurant du remplissage des stockages jugés indispensables, on garantirait durablement la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel sur le territoire français. ces stocks serait du seul ressort du ministre de l'énergie et permettrait d'assurer la continuité de fourniture des consommateurs de gaz en cas de mise en oeuvre du plan d'urgence « gaz » élaboré sur le fondement de l'article 10 du règlement n° 10 du règlement n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010. Ce type de dispositif a déjà fait ses preuves dans d'autres pays européens, comme l'Italie, la Hongrie ou la Pologne, ainsi qu'en France dans un autre domaine relativement similaire, en pétrole. En effet, pour remédier aux conséquences d'une crise d'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers, en provenance en particulier de pays tiers, la France a, comme la majorité des pays industrialisés,

à prévoir, en cas d'insuffisance des capacités souscrites après mise aux enchères, la possibilité d'imposer, en dernier recours, aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires. S'agissant des contraintes imposées aux stockeurs, les notions de stocks stratégiques et de stocks complémentaires sont en réalité très voisines. Elles ne diffèrent que par la possibilité de conserver tout ou partie

manière, pour nous, de tirer les leçons des événements de l'hiver dernier -et repose notamment sur une commercialisation aux enchères des capacités de stockage, afin de restaurer leur compétitivité tout en incitant à proposer des offres optimisées pour satisfaire les besoins des consommateurs. Afin de garantir la constitution, en amont de l'hiver, des stocks de gaz nécessaires au fonctionnement du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement, un « filet de sécurité » est prévu à l'article L. 421-6 en cas de souscription insuffisante au moment des enchères. Les fournisseurs de gaz naturel conservent par ailleurs une obligation d'assurer un approvisionnement continu de leurs clients, y compris dans des conditions froides telles qu'il s'en produit statistiquement une fois tous les cinquante ans. L'ajout de stocks stratégiques en complément de ces dispositifs

souscrit une capacité de stockage d'assurer le remplissage de celle-ci. Le respect de l'obligation de remplissage étant vérifié au 1 novembre, à une date où il n'est plus envisageable de constituer de nouveaux stocks, cette mise en demeure nous paraît inutile. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le respect

le ministre d'État. Cet amendement vise à rendre explicite la couverture des coûts de recherche et développement pour les opérateurs d'infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, comme cela est prévu pour les autres opérateurs régulés.

régulés. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à préciser explicitement que les coûts de recherche et de développement des opérateurs de stockage seront couverts par les tarifs. Cette précision est de nature à rassurer et ne pose pas de difficulté sur le fond, une telle couverture étant déjà prévue pour les autres opérateurs régulés. L'avis est donc favorable.

peuvent comporter », et non plus « comportent », les trois parts mentionnées ici, dont la part proportionnelle à la modulation hivernale ayant vocation à être utilisée pour couvrir le coût du stockage. Les tarifs actuels comportent en effet d'autres termes, qu'il convient de ne pas exclure par une rédaction trop restrictive.

telle qu'elle figurait dans le projet d'habilitation initial. S'il n'y a plus lieu de prévoir une telle réduction pour compenser les effets de la réforme du stockage, dans la mesure où le mécanisme additionnel d'interruptibilité ajouté par la commission des affaires économiques exonérera de fait ces consommateurs de la hausse du tarif qui en aurait résulté, une modulation des tarifs pourrait cependant, de notre point de vue, rester nécessaire dans le cadre de la définition des règles du délestage. Ces règles pourraient en effet conduire à entériner le fait que

l'absence de relations entre le transporteur de gaz, le gestionnaire du réseau et la société filiale qui opère des terminaux,

de la gestion des réseaux. À cette occasion, la France avait obtenu qu'un modèle dit de « gestionnaire de réseau de transport indépendant » puisse être retenu, pour permettre à nos entreprises nationales de rester propriétaires du réseau, à condition que sa gestion soit assurée par une entreprise totalement indépendante. Revenir sur ces règles aujourd'hui pour l'ensemble des gestionnaires de réseaux risquerait de fragiliser ce modèle français, qui plus est pour traiter un cas d'espèce qui relève de la politique d'investissement d'une société particulière. L'avis est défavorable.

La réglementation européenne n'autorise effectivement une entreprise historique verticalement intégrée ayant une activité dans la production et aussi la fourniture de gaz naturel à conserver le contrôle d'un gestionnaire de réseau de transport

est à M. Roland Courteau. La commission des affaires économiques a modifié la rédaction de cet article introduit par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle a notamment étendu l'indemnisation du producteur aux avaries ou aux dysfonctionnements survenant sur l'ensemble du réseau d'évacuation, non pas seulement sur la partie marine. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par les députés en supprimant l'extension au réseau terrestre du régime d'indemnisation pour les parcs d'énergie marine renouvelable, prévu initialement pour couvrir les seuls risques d'avarie sur la partie marine du raccordement. En effet, si la spécificité du milieu marin et les contraintes pesant sur toute opération en mer- aléas météorologiques, disponibilité des matériels et des bateaux -justifient que la collectivité assume le risque représenté par des délais de réparation de plusieurs mois, afin de réduire les coûts liés et le coût final du projet supporté par les consommateurs- c'est l'objet même de la réforme proposée par le Gouvernement et RTE -, il n'en va pas de même pour le réseau terrestre. La partie terrestre du raccordement pour les énergies renouvelables en mer est en effet semblable à tout raccordement de site de production terrestre, techniquement comme en termes de risques d'avarie. Dès lors, comment justifier que les producteurs d'énergie en mer soient automatiquement indemnisés en cas d'avarie sur leur raccordement terrestre, alors qu'aucun autre site de production terrestre ne bénéficierait du même avantage En effet, l'indemnisation des producteurs à terre, toutes énergies confondues, demeurerait subordonnée à la démonstration d'une faute de RTE, conformément aux cahiers des charges du réseau public de transport. En application du principe d'égalité des usagers du service public, une telle différence de traitement doit être justifiée par des critères objectifs, en lien direct avec l'objet de la disposition législative. Les modifications adoptées en commission comportent ainsi un risque sérieux de voir contesté l'ensemble du régime applicable au réseau d'évacuation terrestre,

Tel ne sera pas le cas si le dispositif reste limité à l'indemnisation des avaries sur la partie marine du réseau, ce que justifie pleinement la complexité des réparations en mer et des facteurs exogènes pesant sur celles-ci.

production, et, d'autre part, à l'ensemble du réseau d'évacuation, au lieu de la seule partie marine de ce réseau. Les auteurs de l'amendement centrent leur argumentation sur cette seconde précision et craignent un « risque de contagion à tous les raccordements terrestres ». même sur le respect du principe d'égalité par cette disposition. Je rappellerai que ces modifications sont justifiées par le fait que les conséquences économiques d'une indisponibilité du réseau, qu'elle soit liée à sa partie marine ou à sa partie terrestre, sont identiques pour le producteur. J'ajoute que les risques sur la partie terrestre sont bien mieux maîtrisables- et maîtrisés -par RTE. Ces dérogations ne sauraient par ailleurs servir d'argument aux producteurs d'énergies renouvelables terrestres pour demander à bénéficier d'un régime équivalent, puisque leur justification tient uniquement au fait d'évacuer la production d'installations implantées en mer ; il n'y a donc pas de « risque de contagion Les auteurs de cet amendement n'ignorent pas que les énergies marines renouvelables bénéficient déjà, depuis la loi Autoconsommation, d'un régime dérogatoire du droit commun. Il n'y a pas là de rupture d'égalité puisque l'on traite bien différemment deux situations objectivement différentes, entre les installations terrestres, d'un côté, et les installations marines, de l'autre, l'autre, dont le réseau d'évacuation aboutit nécessairement à terre. C'est par ailleurs la logique même du nouveau système proposé que de « dérisquer » les projets pour faciliter leur réalisation. Nous allons donc au bout de cette logique.

Je rappelle que, dans le nouveau cadre du raccordement des installations d'énergie renouvelable en mer, l'ensemble de ce raccordement est réalisé par le gestionnaire du réseau de transport. Les conséquences d'une défaillance sont les mêmes qu'il s'agisse de la partie marine ou de la partie terrestre.

pour l'évacuation de l'ensemble des sites de production d'électricité terrestre, quels que soient l'énergie concernée, son mode de financement et son amortissement. Imaginons l'incidence d'une telle mesure- parce qu'il y aura bien contagion -pour l'évacuation des sites de

et un plafonnement de l'indemnité peut alors se justifier. Dans d'autres cas, la responsabilité du gestionnaire de réseau sera pleinement engagée et, dans ces conditions, l'indemnité devrait couvrir la totalité du préjudice subi par le producteur. Cet amendement vise donc à supprimer l'introduction d'un plafonnement de l'indemnité dans la loi, pour renvoyer à un

Le nouveau cadre de régulation des raccordements d'éoliennes en mer déroge déjà largement au droit commun dans un sens favorable aux producteurs et contribue à réduire très fortement leurs risques, ce qui devrait d'ailleurs faire baisser le coût global pour la collectivité. Déplafonner totalement ces indemnités remettrait en cause l'équilibre trouvé entre l'intérêt des producteurs et celui des consommateurs, qui me paraît satisfaisant. J'ajoute qu'en intégrant les cas de dysfonctionnements et en visant la totalité du réseau d'évacuation, notre commission a déjà considérablement amélioré le texte du point de vue des producteurs.

Dans le projet de cahier des charges, objet du dialogue concurrentiel actuellement ouvert, il est demandé au lauréat de constituer, au moment de l'attribution du projet, des garanties bancaires qui seront exécutées en cas de défaillance

L'ajout d'une garantie supplémentaire émise par le lauréat afin de garantir les coûts engagés pour le raccordement en cas de défaillance crée une accumulation d'engagements et de risques peu cohérente avec le but visé, à savoir la baisse des prix de l'électricité. Ce risque supplémentaire Ce risque supplémentaire pour le lauréat est par ailleurs difficilement quantifiable par ce dernier, dans la mesure où il n'exerce aucun contrôle sur le programme d'études et de travaux de RTE, et donc sur les coûts internes et externes engagés par le gestionnaire du réseau de transport. Décorréler les travaux de RTE de ceux du lauréat est d'ailleurs l'un des objectifs du nouveau dispositif. de progresser en amont du calendrier du projet, afin de limiter son risque de retard. À titre de comparaison, dans le schéma allemand, dans lequel les risques et les coûts du raccordement sont transférés au gestionnaire de réseau, le lauréat ne fournit aucune garantie spécifique en relation avec cet aspect du projet, la garantie générale constituée par lui au titre de l'appel d'offres étant considérée comme suffisante.

Ces derniers doivent en effet assumer les conséquences financières des coûts supplémentaires qui résulteraient soit de leur initiative, soit de leur défaillance. L'avis est donc défavorable.

base de la solidarité entre territoires urbains et ruraux. Le développement de tels réseaux fragiliserait ainsi la péréquation tarifaire et créerait une rupture d'égalité entre les consommateurs reliés à ces réseaux et les autres. C'est pourquoi ils doivent être limités aux situations strictement nécessaires. Celles-ci sont déjà prises en compte aux articles L. 344-1 et suivants du code de l'énergie relatifs aux réseaux fermés de distribution, qui peuvent répondre, sous conditions, aux situations de ports, d'aéroports, de sites industriels et commerciaux, de bâtiments à usage tertiaire. Ainsi, la création d'une troisième catégorie de réseaux pour des immeubles de bureaux nécessite une analyse de sa compatibilité avec la directive européenne 2009/72/CE du 13 juillet 2009, qui n'en prévoit que deux afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et les droits des consommateurs la catégorie générale, qui comprend en France les réseaux publics exploités par Enedis et les entreprises locales de distribution, et la catégorie des réseaux fermés.

Pour mémoire, les articles L. 315-2 et suivants du code de l'énergie définissent le cadre de l'autoconsommation collective pour les consommateurs raccordés au réseau public. La création de cette nouvelle catégorie mettrait le réseau public au service de l'autoconsommation, aussi bien individuelle que collective. Il est donc proposé de surseoir à la création de cette troisième catégorie de réseaux afin d'en étudier au préalable l'impact sur la péréquation tarifaire les recettes fiscales, la conformité au droit européen et les conditions juridiques, techniques, financières et d'accès au marché de l'électricité applicables à de tels réseaux.

Le texte adopté par notre commission répond aux craintes exprimées par ses auteurs en limitant strictement cette notion aux seuls immeubles de bureaux et aux bâtiments et parties de bâtiments contigus, ce qui préserve la péréquation tarifaire.

unique du bâtiment sans régler le litige pouvant survenir lors de l'aliénation d'une partie de ce dernier. Elle permettra enfin de laisser le libre choix de la norme applicable au réseau intérieur selon que le propriétaire envisage une cession au gestionnaire de réseau ou non. L'amendement n° 84,

le monopole de la distribution publique et la péréquation tarifaire. Au surplus, la rédaction retenue par la commission traite le seul problème identifié à ce jour, c'est-à-dire celui de certains immeubles de bureaux. les mesures prévues au titre des réseaux intérieurs aux immeubles d'habitation et aux bâtiments publics, ainsi qu'aux bâtiments tertiaires ou industriels, sans aucune justification et sans qu'aucune étude d'impact ait été réalisée. précise, en réponse aux auteurs de cet amendement, que la condition de propriété unique du bâtiment n'a pas été ajoutée par notre commission : elle figurait déjà dans le texte adopté par l'Assemblée Notre commission a bien réglé « le litige potentiel survenant lors de l'aliénation d'une partie » du bâtiment : il est prévu que, dans ce cas, le réseau intérieur réintégrera le réseau public de distribution, sous condition de sa remise en état aux frais de son propriétaire. En conséquence, j'émets un avis défavorable

à la maille d'un poste de distribution publique d'électricité. Les projets émergents, actuels ou à venir, révèlent que plusieurs postes publics de transformation d'électricité de moyenne à basse tension sont nécessaires pour mutualiser les effets redistributifs. Par là même, ces équipements induisent une redondance administrative et technique dans le montage des projets. j'attends l'avis de Mme la rapporteur.

est à M. Ronan Dantec. L'obligation d'achat pour les énergies renouvelables est aujourd'hui accessible à des organismes agréés autres que l'opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. mesure concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l'autoconsommation. Toutefois, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, se révèle complexe. Elle souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre, d'un côté, l'opérateur historique les entreprises locales de distribution et, de l'autre, les acteurs agréés, que l'on a acceptés à ce titre. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l'autoconsommation auprès de ses clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut procéder directement. Il doit nécessairement faire intervenir ou une entreprise locale de distribution. Mes chers collègues, afin de simplifier- j'insiste sur ce terme -la gestion des contrats d'obligation d'achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d'exercer librement leur droit à la concurrence- -, ... Ah ! ... dans le cadre de l'obligation d'achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateurs, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l'opérateur historique et de fluidifier le transfert des contrats d'obligation d'achat entre les différents organismes agréés. Au travers de cet amendement, nous vous invitons donc à simplifier cette procédure sur trois points : permettre aux organismes agréés de signer le contrat d'achat initial d'une installation en conséquence, modifier les conditions de cession des contrats en permettant une fluidité entre les acheteurs agréés ; enfin, supprimer la contrainte d'une cession de contrat au 1 janvier de l'année suivante, laquelle n'a pas lieu d'être, notamment au regard des délais d'instruction des demandes. Je précise que ces dispositions ne remettent nullement en cause la solidarité tarifaire entre les territoires.

Revenir dès à présent sur ces modalités me semble très prématuré. Sur le fond, la suppression du guichet unique, proposée cet amendement, conduirait à une hausse des coûts pour les gestionnaires de réseaux, sans que le gain pour ceux-ci soit avéré.

On peut comprendre, et même éprouver l'envie d'élargir le champ des entreprises en mesure de souscrire un contrat d'obligation d'achat. Toutefois, il faut l'admettre, ce sujet paraît assez éloigné des autres dispositions du présent projet de loi ; il mériterait sans doute un débat plus large.

d'informer l'ensemble des consommateurs de la part de biométhane contenue dans le gaz qu'ils consomment. L'article adopté en commission limite cette obligation aux consommateurs souscrivant volontairement une offre verte. Cette disposition semble réductrice et éloignée des exigences de transparence exprimées par les consommateurs. Mes chers collègues, nous vous proposons donc de revenir à la rédaction initiale du présent

la vente n'était pertinente que dans le cadre des offres dites « vertes » de gaz qui comportent une part de biométhane. Compte tenu du faible développement actuel de la filière, cette proportion n'atteint, au mieux, que quelques points

Monsieur le ministre d'État, nous partageons avec vous la nécessité de porter un regard large, transversal et à long terme sur ces sujets intimement liés, à savoir l'énergie, les productions alimentaires, le respect de la biodiversité et les équilibres climatiques. Je proposerai tout à l'heure un amendement visant à mieux prendre en compte le changement d'affectation des terres permettant de produire des agrocarburants, plutôt que de nourrir des humains. Les agrocarburants, il faut le dire, sont en concurrence avec les productions vivrières dans un certain nombre de pays, et ce du fait du scandaleux accaparement des terres, que ce soit par des pays ou par des sociétés multinationales. Ils sont aussi en concurrence avec la forêt primaire, que l'on continue de déforester très souvent pour ces productions.

Peut-on un jour- le plus tôt possible ! -interdire l'incorporation d'agrocarburants de première génération, qui font, eux, directement concurrence aux cultures alimentaires, et n'autoriser que l'incorporation d'agrocarburants de deuxième génération, qui ne consomment que des résidus et des déchets issus de l'agriculture,

les scientifiques estiment que le remplacement des carburants fossiles par les agrocarburants actuels correspondrait au moins à 22 % des productions végétales terrestres, augmentant ainsi de 50 % l'appropriation de cette ressource par l'homme, et contre l'homme, et pourrait compromettre la survie des autres espèces qui en dépendent.

Les biocarburants français et européens subissent une concurrence déloyale des biocarburants importés à double titre. D'une part, les biocarburants importés sont plus facilement l'objet de fraudes aux critères de durabilité, et moins facilement soumis à des contrôles sur place. D'autre part, certains biocarburants importés bénéficient non seulement d'un dumping, mais aussi de subventions qui permettent à leurs exportateurs de les vendre à des prix inférieurs au coût des seules matières premières dans l'Union européenne. Dans ce contexte, une plainte anti-subvention va prochainement être déposée à la Commission européenne pour dénoncer certaines de ces pratiques. Toutefois, le temps que cette plainte aboutisse à des mesures concrètes, l'afflux des biocarburants importés non durables et subventionnés

Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans les installations mises en service après le 1 janvier 2008, l'objet du présent amendement est de mettre en place des mesures provisoires à relever le niveau d'exigence en termes de durabilité- je parle des émissions de CO2 -, le temps que la Commission prenne les mesures appropriées et nécessaires. Le caractère Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d'une part, de lutter contre la concurrence des biocarburants importés

l'amendement n° 76 rectifié . La Commission européenne a décidé de baisser les taxes à l'importation de biocarburants, taxes antidumping, établies en 2013. Cette décision combinée en une nouvelle réglementation en baissant le taux d'incorporation de diester dans la composition du biodiesel que cet article vise à transposer a pour effet de soumettre la filière à une concurrence accrue. Or, tout comme en 2013, cette concurrence est toujours déloyale. Je pense- cela vient d'être dit -notamment aux subventions massives dont bénéficient les biocarburants argentins ou indonésiens par exemple. Certains producteurs eux-mêmes sont épinglés par les « Paradise papers », qui font l'actualité, comme le groupe Louis-Dreyfus. Les acteurs nationaux de la filière sont en train de déposer des recours auprès de la Commission européenne. Je pense également aux problèmes de durabilité que posent ces biocarburants importés et élaborés pour la plupart sur des sites ouverts après 2008. Concrètement, ces amendements doivent permettre de suspendre la décision de la Commission européenne le temps que les recours aboutissent, afin d'éviter des importations que nous jugeons déloyales et litigieuses pendant la durée d'examen du recours. Les enjeux sont importants, avec un impact direct sur l'emploi.

Voilà les premières conséquences de l'annonce, le 13 octobre 2017, par le groupe alimentaire Avril, des mesures de chômage partiel pour 2018 dans les usines de sa filiale Saipol, en raison de la « menace » que fait peser la réouverture du marché européen au biodiesel argentin. Ce dispositif, qui court sur six mois renouvelables à compter de février 2018, concerne environ 250 des 600 salariés de Saipol, répartis dans l'ensemble des cinq usines d'estérification de la filiale en France, dont l'une est située, je le rappelle, à Sète. La raison invoquée est que l'Union européenne a rouvert ses portes, à la fin de septembre 2017, aux importations en provenance d'Argentine, après avoir érigé en 2013 contre les biocarburants en provenance de ce pays une barrière douanière qui a été désavouée par l'Organisation mondiale du commerce. En effet, les subventions permettent aux exportateurs argentins de vendre du biodiesel à un prix inférieur au coût des seules matières premières dans l'Union européenne. L'Association des producteurs de biodiesel européens a annoncé, en septembre 2017, son intention de déposer une plainte auprès de la Commission européenne contre les importations argentines. En l'absence de contre-mesure efficace de l'Union européenne, les conséquences pour cette filiale seraient sans appel, et des centaines d'emplois seraient concernés. Je me réjouis de voir que la prise de conscience est commune, puisque cet amendement, cosigné par des représentants de l'ensemble des groupes de la majorité sénatoriale, est aussi présenté par d'autres groupes de cette assemblée. Étant donné que les biocarburants non durables et subventionnés sont majoritairement produits dans des installations mises en service après le 1 janvier 2008, l'objet de cet amendement est de mettre en place des mesures provisoires visant à relever le niveau d'exigence en termes de durabilité- émissions de CO2 -le temps que la Commission prenne les mesures Le caractère provisoire de cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d'une part, de lutter contre la concurrence des biocarburants importés lorsque celle-ci est déloyale et, d'autre part, de se conformer pleinement au droit de l'Union européenne et de l'Organisation mondiale du commerce.

En septembre dernier, l'Union européenne a pris la décision de réduire significativement les droits antidumping appliqués au biodiesel argentin réalisé à partir de soja. Telle est la concurrence déloyale qui va être installée grâce au gouvernement français, si rien n'est entrepris ! Une hausse Une hausse massive des importations de ce carburant fait craindre des effets désastreux non seulement sur l'environnement, mais aussi sur un secteur de l'économie performant, qui verra ses emplois sacrifiés. Au total, près de 20 000 emplois

puis, demain, indonésien avec l'huile de palme, massivement subventionné par leur pays d'origine et soumis à des critères de durabilité moindres qu'en Europe.

Cet amendement tend à relever le niveau d'exigence en termes de durabilité, c'est-à-dire en termes d'émission de gaz à effet de serre pour tous les biocarburants importés sans exception. Il a pour objet d'éviter à la filière des biocarburants français de se trouver broyée par la concurrence internationale. Cette mesure garantit un juste équilibre entre la nécessité, d'une part, de lutter contre la concurrence des biocarburants importés lorsque celle-ci est déloyale et, d'autre part, de se conformer pleinement au droit de l'Union européenne et de l'OMC.

comme l'ont relevé nos collègues, ce sont plusieurs milliers de tonnes de biocarburants qui vont venir saturer le marché français et évincer la production locale, sans respecter les règles du jeu. D'ores et déjà, une plainte a été déposée auprès de la Commission européenne, mais, avant qu'elle n'aboutisse, la filière pourrait être en très grande difficulté. C'est pourquoi il nous faut agir dès à présent, tout en évaluant les risques juridiques de chacune des solutions proposées. La première série d'amendements- les amendements 13, 40 et 76 rectifié -retiendrait, pour toutes les installations, qu'elles soient françaises, européennes ou d'un autre État tiers, la même date à partir de laquelle les critères de durabilité seraient durcis. Il n'y aurait pas de discrimination selon l'origine des biocarburants, mais on risquerait alors des effets de bord. La seconde série d'amendements- les amendements

La France pourrait cependant faire valoir, d'une part, qu'il s'agit là de répondre en urgence à une pratique anticoncurrentielle dont elle est la victime, et, d'autre part, que la réponse est strictement proportionnée, car limitée dans le temps, jusqu'au 30 juin 2019. Le risque d'une condamnation semblant dès lors mesuré,

qui tendent à modifier les dispositions de la directive de 2015, visent à faire en sorte que toutes les installations mises en service depuis le 1janvier 2008 produisent des biocarburants présentant un niveau de réduction de gaz à effet de serre de 60 % par rapport aux mêmes émissions générées par des carburants fossiles,

41 rectifié et 77 rectifié visent à imposer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus élevé pour les biocarburants produits hors de l'Union européenne que pour ceux qui sont fabriqués à l'intérieur de l'Union européenne. Cette proposition ne pénalisera pas de fait les sites de production française mis en service avant le 5 octobre 2015 et devrait restreindre fortement, selon nous, l'importation du biodiesel argentin. La conformité de cette proposition au droit de l'Organisation mondiale du commerce, il faut bien l'avouer, est en cours d'examen, et les contacts engagés avec la Commission européenne pour le traitement rapide de la plainte déposée par les producteurs de biodiesel

précisément de la filière oléoprotéagineuse, qui a créé 20 000 emplois et qui produit, je le répète, des tourteaux dont nous avons besoin pour l'élevage français.

que la Commission européenne mette en place un système de traçabilité du puits à la roue obligatoire, afin d'éviter les fraudes de la part de ceux qui jouent sur la disparité entre les législations nationales.

M. Guillaume Gontard. Nous proposons cet amendement à l'alinéa 4 de l'article 6 afin de prendre en compte la notion de changement d'affectation des sols indirect et de compléter, ce faisant, la méthodologie d'évaluation des biocarburants. Si l'intention peut paraître louable, l'utilisation des biocarburants soulève des problèmes qu'il nous faut prendre en considération ; notre collègue Joël Labbé vient de le rappeler. En France, quelque 75 % des biocarburants utilisés proviennent de l'huile de palme, dont l'exploitation a des conséquences sur le couvert forestier. Ainsi, le biogazole à base d'huile de palme aurait, selon une étude de la Commission européenne, un impact sur le climat trois fois pire que celui du gazole issu du pétrole. L'évaluation de l'impact environnemental des biocarburants est aujourd'hui incomplète, en particulier parce que sa méthodologie ne prend pas en compte les changements d'affectation des sols indirects. C'est cette lacune que cet amendement

Nous proposons donc d'aller au bout des bases posées par le plan climat, en nous donnant les moyens d'évaluer au plus juste l'impact environnemental de nos pratiques. L'amendement n° 54 rectifié, présenté

envisagée d'une formule qui permettrait de calculer les émissions annualisées résultant de la modification des stocks de carbone au plus près de la réalité. Si une telle formule est adoptée,

le savez, désigne par exemple des matériels agricoles ou des tondeuses à gazon. Or l'Union européenne exige non seulement que les consommateurs soient clairement informés des contraintes d'utilisation des carburants mis en vente, mais aussi qu'une distribution suffisante des carburants compatibles avec tout type de véhicule reste assurée, afin de veiller, en particulier,

catégorie des gazoles ou catégorie des essences. Ce dispositif laisse donc la possibilité à l'arrêté ministériel de préciser les modalités de maintien d'une distribution adaptée au parc de véhicules et n'impose pas directement de contrainte géographique. Les modalités de maintien de la distribution seront à discuter lors de l'élaboration de l'arrêté ministériel. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement

que quelque 28 000 stations-service ont fermé entre 1985 et 2016, et que les 11 000 stations restantes n'assurent déjà plus un maillage optimal du territoire. Tout cela justifie que nous ayons prévu la garantie d'une couverture géographique appropriée, avec une clause de revoyure annuelle.

les mesures fiscales contribuant fortement à la modification des habitudes de consommation des automobilistes. Dans ce contexte, la disparition de la révision annuelle de l'arrêté précisant les modalités du dispositif fragiliserait selon moi la visibilité des distributeurs sur la nécessité du conditionnement au regard de la demande effective. Le Gouvernement fonde son argumentation sur la compatibilité des carburants avec les engins de jardinage, comme les tondeuses

Même si, selon l'Agence européenne de l'environnement, les politiques d'amélioration de la qualité de l'air produisent des résultats tangibles, la pollution de l'air reste un problème majeur. Les trois polluants les plus préoccupants pour la santé

ce sont les particules ultrafines, plus dangereuses encore que les autres et qui conduisent à l'exacerbation des maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Il semblerait que, pour la première fois, des chercheurs aient démontré qu'une hausse de 10 microgrammes

sur la combustion du charbon, si la Pologne et l'Allemagne, qui recourent beaucoup à ce combustible, sont fortement touchées en termes sanitaires,

Selon cette étude, on dénombrerait en 2016 quelque 50 décès liés à l'activité française, mais 460 importés d'Allemagne et 160 de Pologne. Depuis Tchernobyl, nous savons que les frontières n'arrêtent pas les polluants mortels

de la qualité de l'air qui ont reçu le label « ville respirable » en cinq ans, après avoir mis deux ans à échanger avec les services de l'État sur les objectifs et les actions. Il est extrêmement compliqué d'estimer les gains de dioxyde d'azote ou de particules fines que vous ferez avec l'application d'une telle mesure.

Le présent amendement tend à rétablir le caractère obligatoire des mesures visant à réduire l'émission de particules fines dans les périmètres des plans de protection de l'atmosphère, les PPA, qui dépassent les valeurs limites. Ces mesures consistent à favoriser le recours aux énergies et aux technologies les moins émettrices de particules fines et à faciliter le raccordement aux infrastructures gazières publiques et aux réseaux de chaleur existants. Au regard des dépassements fréquents des valeurs limites en matière de particules fines, il est urgent d'agir pour améliorer la qualité de l'air ! Quel

est l'avis du Gouvernement ?

Cet amendement a pour objet, dans un contexte de baisse des dotations de l'État, de permettre aux régions d'outre-mer de bénéficier de ressources fiscales liées à l'exercice de leur compétence de délivrance de titres miniers en mer. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2000, les régions ultramarines de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion sont compétentes pour délivrer les titres miniers en mer de recherche et de production, notamment en matière d'hydrocarbures. Cette compétence, prévue à l'article L. 611-31 du code minier, doit faire l'objet d'un décret d'application, décret toujours non adopté après près de dix-sept ans et malgré deux arrêts du Conseil d'État. Les articles 1519 et 1587 du code général des impôts prévoient actuellement le paiement de redevances au bénéfice des communes et des départements par les explorateurs et les concessionnaires de mines. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux gisements situés en mer au-delà d'un mille marin des lignes de base. Or les titres miniers en mer délivrés par les régions d'outre-mer en vertu de l'article précité du code minier ont vocation à porter sur des périmètres situés largement au-delà d'un mile marin des côtes. Il convient donc d'adapter le code général des impôts à ce type de titres miniers en eau profonde. L'amendement n° 79

Le Gouvernement indiquait dans l'étude d'impact que le décret qui doit préciser les modalités de délivrance de ces titres par les régions d'outre-mer interviendra prochainement. Aussi la commission aimerait-elle connaître l'avis du Gouvernement sur cette question fiscale.

Cet amendement vise à modifier l'article L.631-3 du code de l'énergie relatif aux sanctions applicables pour non-respect des obligations en matière de capacité de transport pour l'approvisionnement stratégique de pétrole brut et de produits pétroliers par voie maritime et à la possibilité pour un assujetti ou un groupement d'assujettis de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture. couverture. Il a pour objet de rééquilibrer le régime actuel, qui ne fait pas de distinction entre le transport de pétrole brut et celui des produits pétroliers dans la détermination du niveau de sanction, une sanction pour un armateur ou un groupement d'armateurs au même titre qu'un assujetti en cas de non-respect de la réglementation. Le dispositif en vigueur fait porter à l'assujetti une responsabilité sur laquelle il n'a pas de prise. Aussi, il est proposé de transférer à l'armateur ou au groupement d'armateurs les obligations de l'assujetti ou du groupement d'assujettis, dès lors qu'un contrat de couverture est signé, et de prévoir pour l'armateur ou le groupement d'armateurs les mêmes sanctions que pour les assujettis en cas de manquement.

pour non-respect des obligations de capacité de transport pour l'approvisionnement en pétrole brut et en produits pétroliers par voie maritime, et de transférer à l'armateur la responsabilité du respect de l'obligation, dès lors qu'un contrat approuvé par l'administration a été signé entre cet armateur et l'assujetti.

qui débutera le 1 janvier 2018. Depuis 2006, ces entreprises ont toujours participé au dispositif des CEE, bien que, dans le cadre de la troisième période d'obligations triennales en cours, les distributeurs de fioul domestique produisent désormais moins de 10 % de leurs obligations. En l'état actuel de la législation, ce secteur d'environ 2 400 entreprises ne pourra plus satisfaire ni répondre aux nouvelles obligations triennales des CEE en raison d'une particularité sectorielle, puisque ce secteur est composé à 90 % de structures de moins de dix salariés, qui délivrent plus de 50 % des volumes de fioul domestique. Cet amendement vise donc à aligner le régime d'obligations portant sur le fioul domestique sur le régime des carburants afin de ne pas isoler des entreprises de la politique de maîtrise de la demande énergétique en France, alors même que le fioul demeure la troisième source d'énergie consommée par les Français

un mécanisme faisant obligation aux vendeurs d'énergies de faire réaliser des économies d'énergies aux consommateurs. Dès l'origine de cette obligation, un dispositif particulier a été reconnu pour le secteur de la distribution du fioul domestique. Ce secteur représentait en effet près de 2 400 entreprises obligées. Au regard des enjeux de la quatrième période d'obligation 2018-2020, qui augmente les objectifs de près de 70 %, il est nécessaire de modifier au plus tôt le régime d'obligations portant sur le fioul domestique. À défaut, ce secteur se trouverait en situation d'échec, du fait de la petite taille des entreprises visées. En effet, 90 % des entreprises de distribution de fioul domestique comptent moins de dix salariés, mais délivrent plus de 50 % des volumes. Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 221-1 du code de l'énergie pour aligner le régime d'obligations portant sur le fioul domestique sur le régime qui prévaut en matière de carburants. La quatrième période débutant au 1janvier 2018, il est proposé que cette modification prenne effet au plus tard le 1 janvier 2019.

est question par des entreprises de plus grande taille, qui sont évidemment mieux à même d'y répondre, à l'instar de ce qui est en vigueur pour les carburants automobiles, tout en préservant, ce qui est important, l'ambition du dispositif des certificats d'économies d'énergie. L'entrée en vigueur différée au 1 janvier 2019 est opportune pour préciser les modalités de transition et préserve le principe de fonctionnement par année civile largement utilisé dans le dispositif. Sans remettre en cause les mérites de ces amendements, ceux-ci tendent à introduire un nouveau sujet dans ce projet de loi. C'est pourquoi

a jugé que cette distinction était sans portée réelle, le projet de loi interdisant en effet toute recherche et exploitation d'hydrocarbures conventionnels et non conventionnels.

le soulignent, le Conseil d'État avait rappelé qu'une telle distinction non seulement n'était pas consensuelle sur un plan technique et scientifique, mais surtout était sans portée réelle et étrangère à l'objectif visé par le projet de loi.

explication de vote. Dans un contexte climatique ô combien inquiétant, alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, tandis que la détresse et la désolation se répandent un peu partout, partout, que le temps joue contre nous et que l'urgence d'agir se fait de plus en plus pressante, voilà que la majorité sénatoriale a pris une décision ne rien faire, pour que rien ne change, c'est-à-dire laisser faire, laisser aller ! Ce n'est pas vrai ! Vous venez de détricoter le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale,

Voilà une belle occasion ratée ! Votre démarche, monsieur le ministre d'État, avait pourtant dès le départ bénéficié du soutien total du groupe socialiste moyennant quelques engagements concernant l'accompagnement des territoires et des entreprises affectés en 2040. Notre groupe était en effet largement ouvert à cette démarche volontariste, qui marquait qui marquait une sorte de passage à l'acte dans la continuité de l'accord de Paris, ainsi qu'une véritable rupture. Enfin, nous allions cesser de reporter les décisions difficiles sur les générations futures

repêchage de plus de quarante demandes de permis de recherche, renforcement des droits acquis et des droits de suite, autant de chevaux de Troie pour ceux qui veulent que rien ne change et partageons même votre lassitude face à une telle mise en cause du texte, et ce en dépit de toutes les argumentations possibles sur le danger d'une telle inertie. Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, par vos rejets successifs de nos amendements, par votre positionnement négatif, qui a

! Deux jours de débats auront suffi pour que les masques tombent. Derrière le consensus de façade sur l'urgence climatique, il existe en réalité une divergence profonde. Bref, deux visions de société s'affrontent. La majorité sénatoriale a ainsi fait le choix de porter des coups à ce projet de loi au nom des droits acquis des titulaires de droits miniers, faisant primer le droit absolu à la rentabilité des intérêts économiques privés, partisans et financiers sur l'urgence environnementale et climatique qui relève de l'intérêt général, ainsi que sur le droit pour tous de vivre dans un environnement sain. Je le dis de nouveau avec force : les plus touchés par le dérèglement climatique sont en premier lieu les plus fragiles et les plus précaires d'entre nous. Au fond, il s'agit du même débat que celui que nous menons autour du CETA, qui privera les États de leur libre arbitre dans les politiques environnementales, notamment, puisque toutes les contraintes pour la liberté des entreprises, même celles qui sont justifiées par la protection de l'environnement ou de la santé publique, pourront être considérées comme illégales par un tribunal d'arbitrage. Pour cette raison, nous continuerons à demander un grand débat public sur la question du CETA et la consultation du peuple par référendum, car c'est de l'urgence de la transition écologique qu'il s'agit.

le signal de l'impuissance de l'État à maîtriser sa politique énergétique et minière, sur le plan tant national qu'international. Or, pour respecter les engagements de l'accord de Paris, quelque 80 % des énergies fossiles doivent rester dans notre sol. C'est une évidence : il n'y a pas d'avenir dans l'exploitation des hydrocarbures ni à court terme ni à long terme. Il faut s'engager clairement et massivement en faveur du développement des énergies renouvelables, de la diversification du mix énergétique, de la formation dans ce secteur et de la mise en place de technologies d'avenir. Pour ce faire, une voie, une seule, nous semble adaptée et pertinente, celle de la création d'un pôle public de l'énergie, dégagé des impératifs financiers dans le cadre d'un marché libéralisé, seul capable d'assumer un service public tourné vers la satisfaction des besoins. Finalement, d'un texte qui comportait des manques, mais qui présentait l'avantage de porter un symbole fort, celui de la fin irréversible de l'exploitation des ressources fossiles à l'horizon 2040, nous arrivons à un texte plat, une loi que

à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels dont nous achevons l'examen présente une saveur particulière. La teneur de nos échanges depuis deux jours en est le témoignage. tour à tour d'affichage, volontariste, puis symbolique, ce projet de loi n'est clairement pas une révolution dans la politique de transition énergétique et de développement durable de notre pays. Les visions proposées par les textes Grenelle I et II, puis le volontarisme affiché dans la signature de l'accord de Paris ont placé la France parmi les nations dans ce domaine. Avec d'autres pays, nous essayons de montrer un autre chemin de développement durable, économique et social. Notre famille politique et le groupe Union Centriste ont toujours suivi et été volontaristes dans ces démarches. Monsieur le ministre d'État, je suis au regret de vous dire que ce projet de loi n'a pas la même épaisseur politique et manque, à notre sens, d'une vision globale. Les sénateurs centristes veillent tout particulièrement à ce que nous nous engagions dans un développement équilibré et à ce que nos grands objectifs en matière d'environnement et de transition énergétique puissent être mis en oeuvre. Ce qui nous intéresse, ce sont les moyens accordés à cette politique et la possibilité de suivre la réalisation de nos objectifs. Puisque ce projet de loi traite notamment des conséquences de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et de la nécessité de réduire notre empreinte carbone, nous attendions plutôt le Gouvernement sur le suivi de ces trajectoires, sur la possibilité d'atteindre nos objectifs nationaux, européens et internationaux, qui sont très ambitieux 80 % des gaz à effet de serre en 2050, avec une étape à 40 % en 2040. Ce qui nous intéresse, monsieur le ministre d'État, ce sont les trajectoires dans les domaines du logement, des transports, de la rénovation thermique, des énergies renouvelables et de la baisse de la consommation énergétique. de ce projet de loi, nous nous sommes demandé pourquoi nous engager dans une sortie complète de la production d'hydrocarbures dans notre pays en 2040, alors que, à cette date, même si nous sommes les meilleurs du monde, nous continuerons d'avoir besoin d'énergies fossiles. nous voulons aussi montrer notre volonté et relever le défi de la lutte contre le réchauffement climatique. De ce fait, sur le fond des sujets, nous vous soutiendrons,

l'espoir de pouvoir coconstruire un texte permettant de mettre la France en position de pionnière dans le débat de la COP23, qui a lieu en ce moment.

et de l'ambition qui le caractérisait à l'origine. C'est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche votera contre ce texte, qui a été dénaturé par le Sénat.

pour ce texte. Nos collègues de l'opposition sénatoriale ont été un peu caricaturaux en voulant faire de l'ensemble de la majorité sénatoriale des climato-sceptiques.

Pour nous, pour notre planète, pour nos enfants, nous nous devions d'être unis et de partager les orientations originelles de ce texte. Comme beaucoup, je suis amer. L'urgence est là, nous devons changer et, pourtant, voilà où nous en sommes : le texte est vidé de sa substance, anéanti. Que croyons-nous ? Que nous pourrons continuer ainsi ? Non, l'ère du pétrole est finie ! Il faut l'admettre et construire une nouvelle ère. Ce texte donnait une direction, une force à notre pays. Aujourd'hui, certains prennent une lourde responsabilité et tournent le dos à la réalité ; c'est pourquoi nous sommes déçus de manquer ce rendez-vous et de devoir voter contre ce texte.

presque deux ans après la COP21, alors que la COP23 débute à Bonn, la situation est alarmante : les États-Unis, deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, cherchent à se retirer de l'accord et les études scientifiques s'accumulent qui mettent en doute la possibilité de respecter le seuil de 2°C. Dans ce contexte difficile, il est impératif de prendre des mesures volontaires et contraignantes, afin de faire respecter nos engagements internationaux sur le climat. Ce projet de loi, visant à mettre fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels en France, aurait pu permettre d'envoyer un signal fort à la communauté internationale. La France aurait pu choisir de s'opposer fermement à l'industrie fossile et aux puissants du du secteur minier. Cela ne sera pas le cas. Notons que, en parallèle de ce volontarisme de façade, le Gouvernement ne semble pas vouloir mettre de frein à la ratification des différents traités de libre-échange transatlantique, pourtant profondément « climaticides ». Les reculs successifs opérés sur ce texte lors de son examen à l'Assemblée nationale et au Sénat ont sérieusement altéré les espoirs placés en lui. Alors que l'urgence climatique est avérée et que tous les signaux sont au rouge, il est regrettable de constater que, sur un sujet si crucial, les avancées ne se font qu'à la marge. Il faut se rendre à l'évidence, les dispositions de ce texte ont une portée trop limitée et les intérêts des industriels du secteur fossile y sont encore trop protégés. Pour ces raisons, je voterai, avec regret, contre ce texte.

La Guyane est devenue en 1964, par la volonté politique du général de Gaulle, une base spatiale. Pour le reste, la Guyane a toujours été administrée de façon un peu chaotique, parce que l'État a surtout voulu y préserver la paix sociale. Aujourd'hui, le résultat est clair.

sous cloche et, aujourd'hui encore, il n'y a pas de développement de notre territoire. Il s'agit donc de volonté politique. La majorité de la population souhaite que nous puissions y voir un peu plus clair, et c'est dans ce sens que nous voterons pour ce texte.

jour d'après ... Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne confiance aujourd'hui. Nous avons travaillé de manière pragmatique sur l'éolien maritime, sur le stockage de gaz, sur les biocarburants.

projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public

Le scrutin est ouvert.

de l'affaiblir, sont recevables individuellement, surtout quand on les traite avec le logiciel du temps présent. ils ne sont pas recevables si l'on se tourne vers l'avenir. Je crains que, ici et ailleurs, nous ne nous entêtions à sacrifier l'avenir au présent. Je suis très inquiet. Pourquoi ? Parce que je sais que l'exercice est difficile. Je sais que l'objectif qui nous est imposé pour éviter que l'avenir ne nous échappe nous obligera à consentir beaucoup plus d'efforts que ceux que ce projet de loi nous demandait. Alors que

probablement des raisons d'être, parce qu'il paraissait assez extraordinaire que l'homme puisse s'être mis dans une telle situation de vulnérabilité. Je comprends qu'il ait fallu que la science